Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a un an, notre pays basculait dans une ère inédite : il était confiné et faisait face à la pandémie. Je voudrais aujourd'hui exprimer la reconnaissance du Sénat à tout le personnel soignant, qui s'est engagé totalement au service de nos compatriotes, et qui

L'implication et le dévouement des professionnels de santé sont exemplaires et nous permettront, je l'espère, d'éviter le pire. En notre nom à tous, je veux leur rendre hommage. Hélas, cette épreuve n'est pas terminée ! Cela renforce encore le sens de cet hommage du Sénat : au-delà du personnel soignant, il s'adresse aux femmes et aux hommes qui, travailleurs de la première ligne, ont assuré l'essentiel dans des moments particulièrement difficiles. C'est grâce à eux que le pays a tenu et qu'il tient encore. C'est grâce à eux que nous continuerons de faire face, forts de nos valeurs de solidarité. Comment ne pas penser à tous nos concitoyens qui ont été victimes de l'épidémie ? Comment ne pas penser à la douleur de leurs proches, à la souffrance de ceux qui n'ont pu entrer en contact

de vous remercier,

Notre peuple souffre, et la maladie frappe, avec plus de 91 000 morts et des milliers de personnes hospitalisées. Elle frappe socialement : la barre des 10 millions de pauvres a été franchie. Elle frappe psychologiquement, particulièrement notre jeunesse. Ce matin, le conseil de défense a décidé de nouvelles mesures. Elles devront être à la hauteur de la nouvelle dégradation de la situation dans nos hôpitaux. En Île-de-France comme dans de nombreuses autres régions, la situation dans les services de réanimation est dramatique, car il n'y a plus de lits pour accueillir des patients en phase critique. Des malades sont transférés, mais les médecins préviennent que la vague est trop forte et que les transferts annoncés ne suffiront pas à l'endiguer. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas ouvert de lits de réanimation ? Vous aviez déclaré péremptoirement : « Il ne suffit pas d'acheter des lits chez Ikea pour ouvrir des places en réa. Hier soir, vous affirmiez encore : « On ne peut pas créer des lits de réanimation supplémentaires d'un claquement de doigts. » Eh oui ! Monsieur le Premier ministre, le temps ne s'est pas suspendu pendant un an. Avec d'autres, nous demandons depuis mars 2020 un changement radical de politique de santé publique, rompant avec la loi de marché. Le 27 août dernier, M. le ministre de la santé annonçait

de ces vaines promesses. Il constate l'affaiblissement de notre système de santé publique et la perte de notre souveraineté sanitaire, puisque nous n'avons pas encore produit notre vaccin. Masques et tests, puis lits et vaccins : notre destin nous échappe, monsieur le Premier ministre. Aussi, quels choix allez-vous effectuer pour ouvrir en urgence, dans les jours à venir, des lits de réanimation ? Allez-vous prendre des dispositions pour sortir les vaccins de la logique du marché, en levant les brevets, et pour accélérer considérablement la réalisation et la production d'un vaccin français ?

! Il ne serait pas raisonnable de laisser accroire que l'on peut, en six mois ou un an, former des personnels aussi spécialisés. ! Que faisons-nous depuis le début de la crise ? Nous reconvertissons d'autres lits, en mobilisant d'autres professionnels hospitaliers, pour accroître nos

santé. Nous sommes donc pleinement mobilisés pour soutenir les établissements hospitaliers et leur personnel, afin de faire face à la résurgence de la pandémie, en même temps que nous travaillons à leur renforcement et à leur transformation structurelle.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons a révélé des fragilités structurelles et un besoin croissant d'infrastructures dans toutes les collectivités. Celles-ci, guidées par des élus locaux engagés, sont naturellement les mieux à même d'identifier et de répondre à ces besoins, comme elles le démontrent quotidiennement sur le terrain.

C'est le cas pour la collectivité territoriale de Guyane, avec laquelle a été signé ce lundi un accord très attendu, que je tiens à saluer. Cet accord territorial de relance pour la période 2021-2022 prévoit un effort à parité de l'État et de la Guyane, à hauteur de 250 millions d'euros, des crédits en supplément de ceux qui ont déjà été octroyés. Cet accord permettra d'accompagner les collectivités et de soutenir leurs projets d'infrastructures. Je pense entre autres, pour les premières opérations arrêtées, au confortement des berges du marché municipal de Grand-Santi, à l'aménagement de la liaison routière Maripasoula-Papaichton et à diverses autres opérations intéressant les collectivités locales. Toutefois, cet accord porte aussi sur le développement économique, de soutenir des projets privés, notamment de production d'électricité fondée sur les énergies renouvelables, de valorisation des produits agricoles, ou encore d'exploitation de nos ressources naturelles. comptes publics, près de six mois après l'annonce de cette nouvelle méthode de coopération entre l'État et les régions, pouvez-vous nous présenter un point d'étape sur la mise en place de ces accords de relance régionaux ?

Avec mes collègues du ministère de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault et Joël Giraud, nous veillons à associer systématiquement les élus à la mise en oeuvre du plan de relance. Les accords régionaux nous le permettent. Une circulaire du Premier ministre nous permet aussi de signer des accords avec des départements et des métropoles ; un accord a notamment été signé avec la métropole de Nantes. Je voudrais enfin saisir cette occasion, monsieur le sénateur, pour rappeler que, dans ce cadre, nous veillons avec beaucoup d'attention sur le partenariat entre le Gouvernement et les collectivités d'outre-mer. Vous avez cité l'accord signé avec la Guyane : vous savez que nous avons veillé à ce que plus de 1,5 milliard d'euros du plan de relance puissent bénéficier aux territoires d'outre-mer.

Un an après, je commencerai mon propos, comme vous l'avez fait, monsieur le président, par une pensée pour les 91 000 disparus, les millions de malades touchés par la covid-19 et les innombrables Françaises et Français fragilisés par cet. Il Il y a un an, devant la situation d'exception qui nous percutait, les hésitations, les urgences, les prises de décisions contradictoires ou encore l'absence de décisions pouvaient faire l'objet d'une forme d'indulgence. Mais aujourd'hui, de situation exceptionnelle en situation exceptionnelle, nous observons une dégradation de la gouvernance de la crise. D'urgence en urgence, c'est la démocratie qui est déstabilisée, ce sont nos libertés qui sont écornées. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin organiser la prise de décision de manière plus démocratique et plus transparente ?

la parfaite transparence des décisions de l'exécutif et de la gestion de cette crise sanitaire, devant la représentation nationale, mais aussi devant l'ensemble du peuple français.

Nous respectons ensuite, me semble-t-il, très scrupuleusement les règles de dévolution des pouvoirs et des compétences applicables dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire, qui nécessite que l'autorité exécutive puisse prendre les décisions qui s'imposent, tout en en rendant compte de façon régulière et diversifiée à la représentation nationale.

-cette après-midi même, après la présente session de questions d'actualité au Gouvernement. Nous n'avons rien à cacher et nous avons même tout à gagner à la transparence, surtout dans l'épreuve collective que traverse notre pays. À À la fin des fins, chacun doit exercer ses responsabilités- la République est ainsi organisée -et le pouvoir exécutif prend les siennes.

pas évoqué le conseil de défense. Depuis un an, ce conseil, dont aucun compte rendu n'est public, est devenu une instance de décision au service d'un pouvoir de plus en plus vertical.

Finalement, le Président de la République a décidé, seul, de faire le pari inverse. Pas de débat parlementaire, pas de discussion organisée ! La parole du Président de la République a suffi, alors que cette décision allait affecter toute la suite de notre stratégie sanitaire, comme nous le voyons aujourd'hui. Pour l'exécutif, le triptyque BFM TV, et ballon d'essai dans les médias suffit à organiser la délibération publique, mais ce n'est pas ainsi que la confiance, si nécessaire pour gagner notre combat contre la maladie, peut se construire. Monsieur le Premier ministre, alors que de nouveaux choix difficiles sont, encore une fois, devant nous, remercie de vous appuyer sur le seul légitime conseil, celui qui représente la Nation : le Parlement Français

En effet, alors que les prestations relatives à ce service sont facturées proportionnellement au tonnage des déchets produits, les recettes destinées à financer ces dépenses sont, pour leur part, soit proportionnelles à la surface des logements assujettis, soit assises sur une redevance au prélèvement difficile, ou sur une taxe ou une redevance qui, hélas, n'a, que trop souvent d'incitative que le nom. Dans ce contexte, les collectivités communiquent de leur mieux, afin d'inviter nos concitoyens, premiers acteurs du dispositif, à mieux trier leurs déchets, de manière à atteindre les objectifs environnementaux ambitieux, mais partagés, qui sont fixés. Toutefois, toute augmentation de cette taxe ou redevance est mal vécue par nos concitoyens, qui ne voient pas leurs efforts récompensés. Cela affecte les plus vertueux d'entre eux : ils risquent d'abandonner le tri, ce qui renchérirait le coût de ce service, avec les dégâts sur l'environnement qu'on imagine. Pour tenter de mieux maîtriser ces coûts, la loi de finances pour 2019 a baissé à 5,5 % le taux de TVA applicable sur l'ensemble des prestations de collectes séparées. Cette baisse de TVA s'applique à compter du 1 janvier de cette année, mais on n'en connaît pas précisément le périmètre.

dans la perspective de mettre en cohérence cette fiscalité avec un objectif : faciliter le tri, aux dépens de l'incinération et de la mise en décharge. C'est ainsi que le Parlement a approuvé, dans cette loi de finances, une augmentation

en 2025. Nous avons souhaité atténuer ce coût pour les collectivités par la mise en place d'une fiscalité plus incitative pour le tri et la collecte des déchets : c'est la baisse à 5,5

Il ne nécessite donc aucun texte d'application, mais nous veillerons, par les instructions données aux services, à ce que ce périmètre soit intégralement respecté et parfaitement appliqué. Le ministère de la transition

tri, et, pour d'autres, de l'incinération ou de la mise en décharge. Pour ce départage des tâches au sein d'un même contrat avec un même prestataire, nous avons encore besoin de quelques semaines de travail, mais je ne manquerai pas de tenir le Sénat informé de la manière dont nous pourrons préciser ces éléments par un texte réglementaire ou par la doctrine.

le 25 janvier dernier, votre administration édictait un arrêté réformant le concours externe du Capes pour différentes matières, dont la langue corse.

À revers de l'histoire, après la réforme délétère du baccalauréat, où les coefficients des langues régionales furent rabotés, décourageant des armées d'élèves et de futurs locuteurs, cette fois-ci, c'est à l'enseignement même du corse que vous vous en preniez en inversant les coefficients de notation, les faisant passer de 7 à 4 pour la langue corse et de 4 à 8 pour le français. En nous proposant un Capes au rabais, vous annihiliez trente années d'efforts et de reconnaissance. Triste ironie, monsieur le ministre, que de si mal réussir la promotion des langues régionales en transformant un Capes monovalent de langue corse en Capes de français option corse suite d'un vote de l'Assemblée de Corse contre cette réforme et de la forte mobilisation des élus de terrain, des syndicats, des étudiants, de l'université et du jury du Capes, il semblerait que votre ministère ait fini par se rendre compte des dommages collatéraux qu'impliquait votre réforme. Ce matin même, Mme la rectrice de l'académie de Corse affirmait que votre ministère, qui avait jusque-là fait l'économie d'un travail important et technique sur les modalités d'organisation du concours, reverrait sa copie concernant le Capes de corse, afin d'en préserver les exigences et les attendus. Monsieur le ministre, nous confirmez-vous que votre ministère reviendra sur l'erreur historique que porte en lui l'arrêté du 25 janvier dernier ? Voilà

En effet, du point de vue des principes, j'ai reconnu à maintes reprises devant la Haute Assemblée ce que dit tout simplement la Constitution : les langues régionales font partie du patrimoine de la France. Oui, nous encourageons l'apprentissage des langues régionales ; personne ne peut chercher à faire croire le contraire.

hebdomadaires en première et six en terminale. Évidemment, cela n'existait pas auparavant. Bien sûr, on doit aussi stimuler la demande des élèves. C'est le cas en Corse. Comme vous le savez, jusqu'à 95 % des élèves y étudient le corse en sixième.

Territoires. Madame la ministre de la culture, je souhaite appeler votre attention sur une situation paradoxale, qui est digne de figurer dans l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de Franz Kafka, où l'absurdité de certaines règles administratives se fait la meilleure ennemie de la liberté d'entreprendre. Nous sommes en pleine crise sanitaire, les salles de concerts sont fermées et les artistes assignés à résidence. La vie culturelle pourrait perdurer de façon dématérialisée, mais les collectivités territoriales et les associations qui organisent des concerts de façon occasionnelle ne peuvent plus passer par l'intermédiaire du guichet unique du spectacle occasionnel, le GUSO. Ce dispositif permet, en temps normal, de simplifier leurs démarches administratives, mais il ne s'applique qu'aux représentations retransmises À titre d'exemple, l'Orchestre symphonique de l'Aube, produit et financé par le département, ne peut plus recevoir son public du fait de la crise sanitaire. Dans l'attente d'une réouverture des salles, un accord a été passé avec une chaîne de télévision locale pour enregistrer, puis rediffuser ses concerts

le département est contraint de conclure en direct près de soixante contrats différents- un par musicien -pour rémunérer ces artistes. je vous sais à l'écoute. Pour sortir de ce cauchemar bureaucratique, accepteriez-vous d'étendre l'éligibilité au GUSO à l'ensemble des concerts et spectacles vivants, avec ou sans public, diffusés en direct ou en différé, sur des chaînes télévisées, internet ou à la radio ? Cette question est d'une grande importance, à la fois pour les musiciens qui sont plongés en apnée dans une année sabbatique forcée et qui se prolonge, et pour l'ensemble de nos compatriotes, qui voient leur accès à la culture entravé. La parole

permet de simplifier les démarches des employeurs. Les captations ne faisaient pas partie des prestations entrant dans le cadre du GUSO,

Monsieur le Premier ministre, comme l'a très bien indiqué tout à l'heure le président du Sénat, Gérard Larcher, cet anniversaire du premier confinement marque aussi symboliquement le surgissement de la pandémie dans notre vie collective. Aujourd'hui, je ne veux pas dresser l'inventaire de ce qui n'a pas marché. Je veux vous parler d'une question majeure, parce que cette épidémie, plus qu'aucune autre crise, a été pour notre pays une épreuve de vérité.

Coupé de toute affection, ce virus nous a arraché des vies. Il nous a peut-être aussi volé une victoire. Sa victoire, c'est notre défaite- une terrible défaite ! -, contre la civilisation,

vous avez fait une description, que je peux partager, des dégâts massifs que cet ennemi invisible a causés non seulement dans nos chairs, mais aussi dans nos valeurs.

Je pense bien sûr, comme vous, à leurs familles, mais aussi à tous ces malades qui ont développé des formes graves, quand ils ont survécu, et qui continuent à porter des stigmates de longue durée, qui affecteront durablement leur vie. durablement leur vie. Les dégâts psychologiques et les conséquences économiques et sociales, comme toujours, ont affecté les plus fragiles et les plus précaires de nos concitoyens.

pour tous les secteurs en souffrance de notre société et de notre économie, des moyens- c'est le fameux « quoi qu'il en coûte » -, pour atténuer les souffrances matérielles et psychiques de nos concitoyens.

On a voulu, sans doute de bonne foi, protéger la vie, mais on a réduit l'existence à sa seule dimension matérielle. En privant ces personnes âgées et ces malades du lien affectif avec leur famille, on les a aussi coupés de leur raison de vivre.

Sa mission était de plancher sur le remboursement de la dette covid. Comment en effet traiter celle-ci ? Connaissant le sérieux et l'expertise de Jean Arthuis, nous devinons qu'il ne sera pas question d'annulation de la dette. Cette idée saugrenue et dangereuse, en effrayant les investisseurs, aliénerait immédiatement notre capacité d'emprunts futurs et nous exposerait à une forte remontée des taux d'intérêt. Comme il n'y a pas d'argent magique, il nous faudra bien rembourser

Le Gouvernement envisage-t-il de cantonner la dette covid, ce qui serait, selon moi, tout sauf une bonne idée ? Enfin, envisagez-vous de sortir, dès 2021, du « quoi qu'il en coûte », comme vous l'avez annoncé, ou comptez-vous attendre 2022, une fois les élections présidentielles

C'est d'autant plus important que nous sommes entrés dans la crise avec une dette plus importante que nombre de nos partenaires européens. Nous avons donc besoin de rétablir progressivement nos comptes publics pour résorber la dette. Cette sortie de crise et la volonté de relancer l'économie devront être évoquées avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre a déjà eu l'occasion, lors de la Conférence du dialogue social, d'inscrire la sortie de crise à l'ordre du jour.

à la proposition de loi organique déposée par Laurent Saint-Martin et Éric Woerth. C'est ensemble que nous pourrons construire une trajectoire de redressement progressif de nos finances publiques.

Quelques voyous ont défié les autorités, parce que celles-ci s'étaient attaquées à leur trafic. Des guets-apens ont été organisés pour piéger les policiers, avec les techniques traditionnelles : tirs de mortier, feux de poubelles et barricades. Face à cette délinquance, des renforts policiers ont été annoncés-

La parole est à M. le garde des sceaux. Les peines planchers, monsieur le sénateur,

la loi prévoit que le conseil des ministres peut révoquer par décret un maire ou ses adjoints. Chaque fois que cette prérogative a été utilisée par le passé- de façon assez rare, fort heureusement -, il a été noté que les faits reprochés privaient l'élu de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

que vous connaissez forcément. Il me semble que le justiciable dont vous parlez a formé un pourvoi en cassation, que la décision, dès lors, n'est pas définitive, et qu'il se débrouille avec sa conscience. Vous demandez à l'exécutif d'intervenir ? Quelle hérésie !

l'absence de mentions sur les étiquettes attestant de l'origine des produits laitiers ne pourra plus être sanctionnée. Néanmoins, la mention de l'origine peut toujours continuer à être indiquée, mais de façon volontaire, par les producteurs.

de l'Union européenne n'a pas jugé le décret de 2016 illégal, elle a énoncé que l'origine du produit ne peut être rendue obligatoire que sous certaines conditions, à savoir la nécessité de justifier un lien entre l'origine ou la provenance du lait. Vous demandez, monsieur le sénateur, quelle sera la réponse du Gouvernement pour ne pas trahir les engagements de la loi Égalim. Mon collègue Julien Denormandie aura l'occasion de formuler très rapidement des propositions, tout particulièrement dans le cadre de l'examen du projet de loi Climat et résilience, de façon à garantir cette possibilité d'étiquetage, et de trouver, avec l'ensemble des parlementaires, les voies et les moyens permettant d'avoir un étiquetage de qualité, qui soit protecteur des consommateurs.

différents orateurs, à savoir le besoin de faire face aux cas de contagion qui, malheureusement, se développent encore plus de nos jours, mais aussi de préparer les conditions permettant, le moment venu, la reprise d'activité pour différents secteurs qui sont aujourd'hui très largement touchés et qui sont en très grande difficulté.

L'avenir est donc largement compromis, et nous manquons de perspective, alors que d'autres pays européens ont exprimé leur ambition de rouvrir et d'ores et déjà élaboré un planning.

Un tel pass sanitaire serait évidemment l'occasion de permettre une reprise graduelle de l'activité dans ces secteurs, comme dans ceux du tourisme, du transport aérien ou de l'hôtellerie-restauration. Ma question est simple : qu'entend faire le Gouvernement pour soutenir ce secteur d'activité ? Souhaite-t-il se saisir du pass sanitaire pour déverrouiller l'économie dans les secteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt ?

vous me permettrez de ne pas entrer dans des considérations qui seraient d'ordre sanitaire ou liées à des problématiques ou des thématiques de circulation et de règles européennes ; cela relève de la compétence d'autres de mes collègues du Gouvernement et de l'autorité du Premier ministre, lequel adapte et prend les décisions en fonction de l'évolution de la situation épidémique.

Nous avons aussi veillé- peut-être y a-t-il encore quelques améliorations à apporter -à ce que l'ensemble des acteurs soit concerné par les dispositifs. Je pense notamment aux salariés, qui peuvent parfois connaître des conditions de vie précaires, avec la multiplication de contrats courts- on parle parfois de « permittents ». Des aides

Nous avons eu l'occasion d'annoncer cette semaine que nous renforcions la prise en charge des coûts fixes, avec un décret, accepté par la Commission européenne, pour les entreprises ayant des chiffres d'affaires importants et caractérisés par des coûts fixes extrêmement lourds.

pour imaginer des reprises d'activité. Les réflexions qu'a engagées Roselyne Bachelot, ministre de la culture, en matière d'expérimentation dans le domaine culturel seront extrêmement précieuses pour accompagner et nourrir d'idées les conditions de reprise d'activité dans le secteur événementiel ou dans le secteur aéronautique. L'essentiel est que les acteurs soient prêts, et c'est ce à quoi nous travaillons.

Le numérique, ce n'est pas que du virtuel. Dans une société qui se numérise toujours plus vite, la résilience informatique de toute l'économie comme de nos services publics devient chaque jour plus essentielle. posent bien entendu la question de la pérennité de nos réseaux, celle de la souveraineté numérique ou de l'hébergement des données, mais aussi celle de la protection contre le piratage et les attaques toujours plus nombreuses. Il est pourtant un risque que nous avons peut-être sous-estimé et que l'incendie des serveurs d'OVH, à Strasbourg, dans la nuit du 9 au 10 mars dernier, vient de mettre en évidence. Cet événement a montré que les atteintes physiques représentaient aussi une menace bien réelle pour nos services virtuels. Ces risques appellent à la nécessaire vigilance autour de tous nos outils informatiques.

Et n'essayez pas de prévenir le régulateur sur l'atteinte des réseaux de communication sur le site « https://jalerte.arcep.fr » : lui-même est toujours inaccessible une semaine après cet incendie L'absence de redondance réelle des données des sites et applications, d'une part, et de plans de reprise d'activité, d'autre part, n'est assurément pas isolée. Les téléservices publics, les données de nos territoires comme celles de nos concitoyens ne méritent-ils pas un coffre-fort numérique plus sûr ? Le numérique est une chance, mais aussi un risque. Il est de notre responsabilité que nos sociétés ne soient plus des colosses aux pieds de silicium. Monsieur le ministre, quelles actions comptez-vous mettre en oeuvre pour garantir que pareil accident ne provoque plus l'arrêt, même temporaire, de nos services les plus essentiels et que l'informatique en nuage ne parte plus en fumée

tout d'abord à vous rassurer : mon collègue Cédric O, immédiatement informé de ce sinistre, a pris tous les renseignements et toutes les précautions nécessaires. Ainsi, pour les principales données de l'État et pour ses réseaux les plus stratégiques, nous gardons une capacité à opérer directement, et le recours à des solutions de stockage en ne nous a pas empêchés de préserver et de dupliquer un certain nombre de données et de faire en sorte que nos bases de données soient parfaitement protégées.

Cela montre le niveau de préparation et de protection des services de l'État. Reste que, je le répète, cet incendie doit permettre une revue de l'ensemble des paramètres, être l'occasion de faire preuve de précaution et inciter l'ensemble des acteurs, pas seulement l'État, à développer des solutions

pas, l'ensemble de ses systèmes, pour servir ses clients et assurer ainsi son rôle de prestataire. L'alerte que nous avons connue est importante ; nous devons y veiller. Mais aujourd'hui, je tiens à être rassurant sur les conséquences que cela aurait pu avoir pour l'État et son fonctionnement.

Or, parmi ces mutations, la dévitalisation de nos territoires ruraux s'amplifie. L'un des exemples les plus emblématiques en est le risque de disparition des derniers commerces de proximité en milieu rural, pour le maintien desquels les élus se sont beaucoup mobilisés, en amenant en amenant leurs communes à devenir propriétaires des murs ou en accordant des exonérations. Rappelons que l'une des particularités de ces petits commerces tient au fait que de multiples activités sont exercées dans un même lieu, avec un café proposant parfois une restauration légère, une épicerie ou un dépôt de pain ou de gaz. Leur viabilité économique, fondée sur la contribution de chacune de ces activités, crise, la fermeture de la partie bar et de la petite restauration ne constitue pas l'activité principale et n'entraîne pas une baisse du chiffre d'affaires supérieure aux 50 % nécessaires à l'ouverture des droits au fonds de solidarité, met en péril économique ces petits commerces essentiels en milieu rural. En effet, comme chacun le sait, c'est la marge sur ces activités de bar et de restauration, largement supérieure à celle des autres activités, qui fait vivre l'entreprise. Monsieur le ministre, devant l'urgence, le Gouvernement envisage-t-il un élargissement des conditions mentionnées au décret du 8 février 2021 donnant accès au fonds de solidarité pour ces petits commerces ? Envisage-t-il, au contraire, une mesure particulière de soutien aux derniers commerces de proximité en milieu rural, afin d'éviter un réel désastre, mettant en péril la vitalité de nos espaces ruraux

dont l'activité peut majoritairement ne pas faire l'objet d'une mesure de restriction et qui n'ont donc pas accès automatiquement aux dispositifs d'aide, notamment au fonds de solidarité, alors même que l'activité considérée comme minoritaire dans le chiffre d'affaires est celle qui peut susciter la marge plus importante, donc la plus grande capacité à vivre. C'est le cas des fermes-auberges et des fermes-restaurants, comme d'un ensemble de petits commerces, souvent logés dans des bâtiments qui appartiennent aux communes et qui ont à la fois une activité d'épicerie, une activité de restauration, ou encore une activité de distribution de presse. de presse. Je vous indique les deux réponses que nous avons d'ores et déjà apportées, et ce sur quoi nous travaillons. La première réponse que nous avons apportée est de faire en sorte que, chaque fois qu'un cas particulier est soumis à notre administration, nous fassions procéder à un examen au cas par cas, de manière à débloquer des situations.

d'inscription ne relève pas de l'éligibilité ou des secteurs S1 et S1 , parce que nous avons tenu compte de l'activité majoritaire exercée. Si nous devons aller un peu plus loin, nous ne sommes pas convaincus que l'extension du fonds de solidarité soit la solution : cela provoquerait malheureusement des effets d'aubaine. Nous cherchons actuellement une solution pour mieux couvrir ces commerces dits « de multi-activités ». Enfin, monsieur le sénateur, votre question est aussi l'occasion pour moi de rappeler devant le Sénat que, aujourd'hui, le fonds de solidarité permet, depuis le début de la crise, d'aider plus de 2 millions d'entreprises,

Un parlement dissous, des morts par centaines, des tortures, des milliers d'arrestations, la loi martiale proclamée, la peine de mort rétablie, l'économie à l'arrêt, la famine qui s'installe, les ONG mises en cause, les entrepôts attaqués et même les pagodes pillées par l'armée

démocratie, ou LND, gagnent plus de 83 % des voix lors des dernières élections législatives ! Aung San Suu Kyi est aujourd'hui au secret. Même ses enfants n'ont aucune nouvelle d'elle, et la fuite en avant continue, la jante osant même l'accuser, ainsi que le docteur Sasa, son représentant à l'ONU, de trahison et de corruption, un mandat d'arrêt international ayant été émis ce matin même contre celui-ci. Face à cette dictature honnie, le mouvement de désobéissance civile unit tous les Birmans, de toutes classes sociales religions et ethnies, y compris, bien sûr, les Rohingyas. Monsieur le ministre, notre ambassade à Rangoon accomplit un travail remarquable, que je tiens à souligner, mais il faut aujourd'hui aller au-delà des déclarations d'inquiétude ou de condamnation. Les sanctions ciblées de l'Union européenne ne seront utiles que si elles englobent toute la famille des dirigeants, notamment leurs enfants. De même, les Birmans espèrent la reconnaissance par la France du CRPH, le gouvernement parallèle issu des urnes. La France a une responsabilité historique. Elle se doit d'encourager le valeureux peuple birman en lutte contre une dictature mafieuse. Elle se doit de montrer au monde qu'elle reste fidèle à ses valeurs de liberté et de droits de l'homme, en entraînant les autres pays à faire de même. Monsieur le ministre, comment convaincre l'Asean, l'Association de sortir de leur neutralité pour s'engager à nos côtés et aux côtés des Birmans ? Et que pouvez-vous nous dire du dialogue avec le CRPH pour mettre fin à une guerre civile de plus en plus meurtrière ?

En outre, nous continuons à suivre de près toutes les ONG qui travaillent en Birmanie, nous maintenons notre aide humanitaire et nous soutenons

de ces événements sportifs, les jeux Olympiques, les JO. C'est une grande chance pour notre pays, pour son rayonnement, mais aussi pour son économie. La seule Coupe du monde de rugby devrait attirer 600 000 visiteurs étrangers, au fort pouvoir d'achat. Selon le comité d'organisation, l'événement pourrait rapporter 3,4 milliards d'euros à notre pays, créer 17 000 emplois, notamment 3 000 apprentis accueillis au sein du comité d'organisation, et générer 119 millions d'euros de taxes additionnelles. pour avoir lieu et se dérouler dans de bonnes conditions, les grands événements sportifs exigent une préparation à la mesure de l'enjeu ; en particulier, les jeux Olympiques réclament, eux, d'importants investissements. la rénovation du Grand Palais, qui doit accueillir les épreuves de judo et d'escrime, vient seulement de débuter. Il faut encore construire le village et la piscine olympiques. En outre, les infrastructures de transport ont pris un retard considérable. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur la préparation de ces grands événements sportifs ? Serons-nous dans les temps, en particulier pour les JO ? Le Japon a dû décaler ses jeux Olympiques d'un an : ne risquons-nous pas d'être contraints de faire de même

Nous avons aussi aidé les organisateurs de différentes façons, en particulier avec le ministère des affaires étrangères, pour permettre que des athlètes internationaux puissent venir. Nous avons aussi travaillé avec le ministère de l'économie pour que les organisateurs puissent bénéficier des soutiens qui valent pour tous les acteurs économiques, mais aussi de mesures particulières, que le Président de la République a fixées lui-même. Je pense en particulier aux compensations de billetterie pour plus de 100 millions d'euros qui ont été décidées voilà quelques mois pour les organisateurs d'événements sportifs.

travaillent à l'organisation. Nous sommes dans les temps ; le compte à rebours est respecté. Cela suppose bien sûr un véritable sens de l'adaptation et une très bonne coopération entre le ministère et l'ensemble des organisateurs. Bien entendu, nous en rendrons compte régulièrement devant la Haute Assemblée.

Elles ont eu respectivement jusqu'à 6 000 et 2 900 emplois. Toutefois, en raison de diverses réorganisations et surtout de la politique de remplacement du diesel par des moteurs électriques, elles n'en ont plus que 3 000 et 1 300. En effet, même lorsque les moteurs électriques sont assemblés en France, la plupart de leurs composants sont directement importés de Chine. S'y ajoute le transfert de plusieurs lignes de production dans d'autres pays européens, le dernier en date étant celui de la nouvelle génération de moteurs turbo à essence, que le président Hollande était venu solennellement inaugurer à Trémery, en 2017. Quatre ans après, il ne reste plus rien : toute la chaîne a été démontée et transférée en Pologne Monsieur le ministre, est-ce cela la politique industrielle de la France ? N'aurait-il pas été plus intelligent d'organiser un recul moins brutal du diesel ? Une fois que l'essentiel du parc automobile aura été électrifié, l'État sera obligé de retrouver des recettes fiscales, en taxant à leur tour les véhicules électriques. Cela prouvera alors que leur compétitivité économique est aujourd'hui complètement artificielle : non seulement leur achat est largement subventionné, mais ces véhicules ne supportent pour l'instant aucune taxe sur le carburant. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour éviter la disparition des deux usines de Trémery et de Metz, qui ont été le fleuron de la conversion industrielle de la Lorraine dans les années 1970 et 1980 ?

Merci, monsieur le président ! Monsieur le sénateur Masson, votre question permet tout d'abord de rappeler l'empreinte historique de l'industrie automobile en Moselle. Vous avez évoqué tout particulièrement le devenir des sites de Trémery et de Metz, qui tous deux appartiennent au groupe PSA, désormais groupe Stellantis après sa fusion avec Fiat et Chrysler. Le site de Trémery fabrique des moteurs diesel, vous l'avez dit ; celui de Metz produit des boîtes manuelles. Nous savons que la conversion progressive du parc automobile et la sortie des énergies fossiles sont plutôt de nature à entraîner une baisse de cette activité, tant des moteurs diesel que des boîtes manuelles, puisque l'essentiel des véhicules hybrides ou électriques a des boîtes de vitesses automatiques. Dans le cadre du plan de relance pour la filière automobile, le groupe PSA, désormais Stellantis, a pris un certain nombre d'engagements, notamment pour reconvertir vers l'électrification la totalité de ses sites de production de chaînes de traction des véhicules. C'est dans ce cadre qu'ont été annoncés deux investissements : un investissement de 60 millions d'euros sur le site de Metz, pour passer de la production de boîtes de vitesses manuelles à la production de boîtes de vitesses automatiques, et un investissement de 140 millions d'euros sur le site de Trémery, pour passer de la production de moteurs diesel à des moteurs électriques.

vers les moteurs électriques ou les boîtes de vitesses automatiques soit la plus protectrice possible de l'emploi. Nous y travaillons avec le groupe Stellantis et nous saurons évidemment rappeler à ce dernier les engagements qui ont été pris, même si, aujourd'hui, nous constatons qu'il les tient et met en oeuvre les décisions qu'il nous avait annoncées. Plus largement, dans le cadre du plan de relance, nous avons la conviction que la reconquête d'une forme de souveraineté industrielle est une priorité majeure. Nous devons faire en sorte de relocaliser des activités et d'accompagner l'innovation, pour sécuriser et stabiliser les emplois industriels, qui sont producteurs de richesse sur notre territoire.

Et alors que l'on en a retrouvé très peu, on fait disparaître ces emplois sans les remplacer ! Ce que je mets en cause, c'est l'absence de conscience du Gouvernement sur la nécessité de compenser les emplois l'on est en train de supprimer par centaines et par milliers sur les sites de Trémery et de Metz.

a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 19 voix pour, aucune voix contre -à la nomination de Mme Florence Peybernes à la présidence du Haut Conseil du commissariat aux comptes.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 L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur ce projet de loi,

Cet amendement vise à compléter le dispositif de mutualisation des services de police municipale en ouvrant la possibilité d'une mise à disposition, pour une commune concernée, d'un ou de plusieurs policiers municipaux relevant du même établissement public de Cette disposition doit permettre à la police municipale de continuer à exercer ses missions en cas d'empêchement, accident ou maladie d'un de ses membres, surtout dans les petites unités de police municipale de deux ou trois agents.

à M. Alain Richard. C'est un sujet sur lequel il faut que nous adoptions une position, et je sais que les avis sont partagés. Il existe une certaine tension, pour ne pas dire une fièvre, sur le marché du travail en ce qui concerne les policiers municipaux. Les recrutements sont difficiles et les besoins des communes souvent intenses. Par conséquent, entre employeurs naturellement tous de bonne foi et de bonne compagnie, nous ne nous faisons pas toujours de très bonnes manières

du sénateur Richard, évoquer la question très importante des polices municipales, de leur recrutement et du mercato, si vous me permettez cette image, qui se produit, notamment lorsque les mairies prennent le soin de recruter et de former ces policiers municipaux. De très nombreux élus, au début en Île-de-France, désormais partout sur le territoire national, évoquent ce mercato, notamment le fait qu'une fois formés ces policiers municipaux quittent le territoire de la commune. Ce n'est pas simplement parce qu'il y aurait ici une police municipale armée et là une police municipale non armée, mais d'abord parce que le statut de la fonction publique empêche localement de verser des primes identiques aux autres fonctionnaires de statut de fonction publique territoriale. Par ailleurs, c'est souvent par les heures supplémentaires, chacun le sait, que l'on offre un certain nombre d'avantages. On provoque ainsi une concurrence assez injuste entre collectivités

avons beaucoup de remontées de la part des maires -, notamment pour les communes les moins attractives et les plus petites, et il risquait d'accroître encore leurs difficultés. Il n'y a pas de pénurie de l'offre sur le marché des policiers municipaux. Le cas de Paris mis à part, plus de 700 policiers municipaux sont inscrits sur les listes d'aptitude et sont en attente d'un poste. Parmi eux, 450 sont en recherche depuis plus d'un an. Une obligation de servir la commune pendant une durée longue combinée à un risque financier pesant sur les agents risquerait donc d'accroître la tendance de ces derniers à attendre une meilleure occasion. Le droit de la fonction publique territoriale prévoit par ailleurs déjà que, en cas de mutation de l'agent dans les trois ans qui suivent sa titularisation, la commune ou l'EPCI d'accueil doit verser à la commune d'origine une indemnité correspondant au montant de la rémunération perçue par l'agent. S'il n'y a pas d'accord sur le montant de l'indemnité, la collectivité ou l'établissement public rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité d'origine. Nous avons donc estimé que le droit en vigueur était équilibré

La personne choisit de passer ce concours et, à ce titre, acquiert une formation qualifiante importante. Évidemment, une fois qualifiée, cette personne est particulièrement concurrentielle sur le marché du travail, notamment dans le privé. Elle doit donc à l'État

Dans notre territoire de la métropole lilloise, monsieur le rapporteur, il n'est pas si compliqué de changer d'employeur, d'être policier municipal à Roubaix ou à Lille, lorsqu'on est policier municipal à Tourcoing.

appartenant à un même département ou à un département limitrophe aux seuls cas de catastrophe naturelle ou technologique. Il est prévu que cette faculté soit limitée dans le temps et exclusivement en matière de police administrative. En conséquence, l'arrêté préfectoral qui en détermine l'application doit impérativement mentionner la durée de cette application exceptionnelle. Quel est l'avis de la commission ?

pour sécuriser des événements festifs, des manifestations exceptionnelles ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique. À ce jour, la mise en commun de policiers municipaux est régie par deux articles du code de la sécurité intérieure, l'article L. 512-3, qui permet aux communes limitrophes ou appartenant à un même EPCI de mutualiser sur le territoire d'une ou de plusieurs d'entre elles, pour un délai déterminé, tout ou une partie des moyens des effectifs de leurs services de police municipale.

Toutefois, une telle possibilité s'exerce exclusivement en matière de police administrative et ne concerne que les policiers municipaux. Or, dans la ruralité, nombre de communes ne disposent que de gardes champêtres. Cet amendement vise donc à permettre à une commune de mettre son garde champêtre à disposition d'une autre au sein de l'EPCI. Quel

La commission des lois a prévu la mise en place de brigades cynophiles dans le cadre d'une police intercommunale sur décision conjointe du président de l'EPCI et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés. Cette méthode consensuelle inspire le présent amendement, qui vise une délibération du conseil municipal pour la création d'une brigade cynophile dans une commune.

une fin de service ordinaire ou une fin de service anticipée, à l'issue de la période active, afin d'envisager son placement dans les meilleures conditions, dès lors qu'il est en parfaite santé et ne présente aucun caractère dangereux. Il s'agit simplement de se montrer soucieux du bien-être de ces chiens, une fois ceux-ci réformés.

municipales, la CCPM, de décider, sur proposition du maire, du président d'EPCI, du préfet ou du procureur de la République, de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale par un service d'inspection générale de l'État. Le Gouvernement propose de supprimer l'avis préalable de la CCPM. Selon lui, le fait que celle-ci ne se réunisse qu'une fois par an en moyenne diffère les déclenchements d'éventuelles vérifications. En outre, la commission aurait davantage vocation à traiter des enjeux nationaux, plutôt que des situations locales.

maires et représentants syndicaux. Il nous semblerait plus approprié de corriger les problèmes relevés par la Cour des comptes, qui a constaté le défaut de communication sur les travaux de la commission, ainsi que l'irrégularité de ses réunions, afin d'en recentrer les travaux sur les seules questions opérationnelles. La commission des lois s'est engagée dans cette voie en adoptant l'article 6 6 B, issu d'un amendement déposé sur l'initiative de notre collègue Françoise Gatel. Dans cette perspective, le maintien de l'avis de la CCPM est justifié, ce qui nous amène à demander la suppression de l'article 6 . Quel est l'avis de la

tous les conventions de coordination qui existent entre les polices municipales et le commissariat ou l'unité de gendarmerie du secteur. C'est une formule tout à fait logique. En même temps, nous savons que, globalement, ces conventions sont

pour de petites interventions est un dialogue entre le maire, avec le policier principal à ses côtés, et l'adjudant de gendarmerie ou le chef de brigade,

La commission des lois rend obligatoires les conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité intérieure pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service de police municipale. Aujourd'hui, elles ne sont obligatoires qu'à partir de la présence de trois agents dans le service. On peut s'interroger sur la portée et l'intérêt d'une mesure, qui va entraîner une certaine rigidité pour les petites communes, d'autant que l'article 6 A 6 A renforce le contenu des conventions, en prévoyant la réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles les communes sont confrontées. Quoi qu'il en soit, dans le contexte de l'expérimentation que la proposition de loi envisage de mettre en place, il convient de rappeler que l'exercice des responsabilités doit être partagé et non confondu. Les forces de sécurité intérieure de l'État constituent l'outil principal de répression des crimes et délits et s'inscrivent dans la phase judiciaire du traitement de ces infractions plaintes, traitement des informations à caractère judiciaire, conduite des investigations, etc. La police municipale constitue l'outil principal de la mise en oeuvre de la politique de prévention de la délinquance décidée par le maire ou le président de l'EPCI.

en raison de la singularité du lien unissant le maire à sa police municipale et du rôle particulier accordé au maire en matière de sécurité publique.

et, de fait, prévoir une composition spécifique lorsque cette commission est réunie en formation de contrôle, avec le Défenseur des droits et un magistrat chargé de la présider. Notre

M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à permettre à des agents de la fonction publique territoriale des catégories A et B de bénéficier d'une assermentation spécifique et de pouvoir ainsi exercer en tant que gardes champêtres. Une telle évolution permet de compléter le cadre d'emploi de catégorie C existant actuellement sans en créer de nouveaux. Cette solution existe déjà pour les gardes particuliers et évite une complexification des grilles indiciaires, déjà très nombreuses.

comme les bois, les forêts et les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du ou des propriétaires concernés, et après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer. L'article, introduit par l'Assemblée nationale,

que la captation d'images, que ce soit au moyen d'un appareil photographique ou d'une caméra, est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Or celui-ci est protégé tant par la Constitution que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu du reste du texte, notamment

après autorisation du procureur et des propriétaires pour arriver à identifier des auteurs de délits, me paraît tout à fait exagérée. Les gardes champêtres sont en première ligne dans nos territoires pour constater certaines infractions, notamment environnementales. Nous devons leur donner les moyens de le faire Quel est l'avis de la commission ?

en séance ... L'amendement n° 3 rectifié est un amendement de cohérence. En effet, depuis le 3 novembre 2017, les gardes champêtres sont compétents en matière de sécurité routière. Toutefois, la législation ne prend pas en compte l'ensemble des procédures et handicape au quotidien ces agents dans leurs missions. Par exemple, le garde champêtre peut immobiliser un véhicule pour défaut de contrôle technique, mais il n'a pas la compétence de le mettre en fourrière. Il doit demander à un officier de police judiciaire. Or enlever un véhicule n'est pas une priorité quand on connaît la masse de travail abattu et les zones géographiques de compétence des groupements de gendarmerie.

Pourquoi les gardes champêtres ne peuvent-ils pas mener des auditions libres aujourd'hui ? Ils peuvent le faire quand ils constatent des infractions au code de l'environnement, ce qui est dans leur coeur de métier. les policiers municipaux, eux, ne peuvent pas bénéficier d'une telle prérogative, même lorsqu'ils sont compétents pour verbaliser des infractions au code de l'environnement.

Quand un garde champêtre a besoin, par exemple, de recueillir le témoignage d'un agriculteur, ce dernier n'est pas toujours disponible et peut venir un jour ou deux plus tard. Cinq jours, c'est donc peu pour recueillir l'ensemble des éléments d'enquête. C'est aussi insuffisant pour décharger significativement les gendarmes. Il convient donc de fixer le délai des cinq jours qui suivent la clôture des faits pour donner pleinement les moyens aux gardes champêtres de leurs compétences, comme c'est dans le cas du code de l'environnement.

mette de côté leur profession, alors qu'ils contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux. Au nombre de 900 aujourd'hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité au coeur de nos territoires, notamment dans les plus reculés Sans nier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale dans certains endroits isolés, notons que les gardes champêtres constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.

a indiqué ceci : « Le placement d'un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de police municipale ou occupant ces fonctions, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions » Il ajoutait : « Si les gardes champêtres ne disposent pas du pouvoir de prescrire les mises en fourrière, ils peuvent cependant pleinement participer à la mise en fourrière d'un véhicule à travers la réalisation de certaines tâches matérielles liées à la procédure, dans le cas où ils sont placés sous l'autorité

Leur action est toutefois limitée à ces tâches matérielles, telles que la désignation de la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule ou la réalisation de la fiche descriptive dressant un état sommaire du véhicule

Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres d'exercer les prérogatives prévues à l'article 28 du code de procédure pénale, qui octroie aux fonctionnaires la possibilité d'appliquer l'article 61-1 dudit code, permettant la conduite d'auditions libres, dès lors qu'il existe à l'égard d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Je tiens à souligner que, en vertu du code de procédure pénale, et par un renvoi au code de l'environnement, les gardes champêtres ont d'ores et déjà la possibilité de recueillir sur convocation ou sur place les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Malheureusement, les auditions qu'ils mènent souffrent de l'absence de ce renvoi à l'article 61-1 du code de procédure pénale, car, en cas de contestation de la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner

Mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de bon sens, qui apporte une sécurité législative aux missions des gardes champêtres en faisant coïncider la loi avec leur mission de sécurité publique. Étendre formellement et clairement aux procédures diligentées par les gardes champêtres les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale relative à l'audition libre d'une personne suspectée garantit que ces fonctionnaires pourront effectuer sereinement leur mission.

C'est la raison de cet amendement de repli, qui ouvre le débat sur la création d'une instance de contrôle du continuum de sécurité que ce texte entend mettre en oeuvre. Une instance indépendante doit pouvoir contester l'intervention des acteurs de la sécurité publique dans sa globalité.

Il s'agit de permettre aux polices municipales d'intervenir, dans le cadre du code de la route, avec ce que l'on appelle des «

doivent pouvoir faire arrêter les véhicules. Aujourd'hui, les forces de sécurité intérieure ont la possibilité d'utiliser ces fameux « sticks », que l'on place devant le véhicule avant qu'il ne redémarre, pour crever les pneus si jamais le conducteur refuse le contrôle.

Nous avions décidé, dans l'article 60 de la loi de transformation de la fonction publique, de permettre aux anciens policiers nationaux et gendarmes de suivre une formation initiale allégée.

Malheureusement, les élus n'ont bien souvent pas connaissance de cette possibilité. Ils se heurtent également à un obstacle pratique, à savoir l'approvisionnement en carnets à souche. à souche. Les plus petites communes ne disposent pas non plus des outils permettant le relevé de l'amende forfaitaire par procès-verbal électronique.

tiennent de la loi, leur donne compétence pour constater toute infraction à la loi pénale par procès-verbal, rassembler des preuves, recevoir les plaintes et prêter assistance à toute réquisition judiciaire, dans les limites territoriales de leur commune. Une réponse ministérielle

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Une première solution serait d'augmenter considérablement les moyens consacrés à leur formation, afin qu'ils puissent exercer l'ensemble de leurs missions dans des conditions convenables. Néanmoins, à défaut d'y parvenir, il nous paraît nécessaire de supprimer certaines de leurs compétences et de recentrer exclusivement autour du contrôle du stationnement et de l'accueil en mairie ou dans les services de police municipale, afin qu'ils ne soient plus exposés inutilement et mobilisés à mauvais escient. L'amendement Brigitte Micouleau. La question de la propreté de nos villes et métropoles se pose de plus en plus, alors même que les incivilités ne cessent d'augmenter

ASVP, aux agents assermentés devant le tribunal de grande instance et aux agents spécialement commissionnés par le maire de verbaliser par contraventions électroniques les infractions liées à la propreté.

le statut des transporteurs de fonds est difficilement applicable à des agents qui effectuent de la maintenance purement technique- je pense notamment à l'obligation d'être armé ou de porter un uniforme.

qui serait soumise au code de la sécurité intérieure, mais qui ne concernerait que la maintenance des automates bancaires. Les agents devraient évidemment être titulaires d'une autorisation d'exercer

Quel est l'avis de la commission ? des prestataires d'automates bancaires. Il s'agit de soumettre les salariés chargés de la maintenance et de la gestion des automates bancaires- en d'autres termes les distributeurs de billets -aux règles applicables aux agents privés de sécurité. Il existe des liens entre la gestion de ces automates et l'activité de transport de fonds, qui est déjà régie par le code de la sécurité intérieure. Un transporteur de fonds qui achemine des billets pour recharger un distributeur est couvert par ce code. Il me semble cependant qu'il existe aussi des différences notables entre ces métiers et ceux de la sécurité. Assurer la maintenance d'un DAB tombé en panne est un métier technique d'une activité de sécurité, même s'il faut bien évidemment s'assurer de la probité du salarié. Je note d'ailleurs que l'amendement vise à mettre en place deux régimes juridiques différents selon que le salarié est ou non en présence de fonds, ce qui n'est pas un gage de simplification. J'observe aussi que l'amendement a pour objet de déroger à l'un des principes essentiels

qui s'applique aux activités privées de sécurité ne fait pas obstacle à la création de filiales dédiées par les constructeurs d'automates ou par les banques, s'ils souhaitent exercer cette activité. Enfin, plusieurs dispositions de

Avec ces dispositions, les 165 000 agents de sécurité privée- un chiffre à comparer aux 21 500 agents de la police municipale ! -sont explicitement intégrés à la politique de sécurité publique. Notre groupe conteste d'emblée cette forme d'externalisation de l'un des piliers de la République, c'est-à-dire les forces de sécurité, vers le secteur marchand. Nous pensons que c'est un aveu d'échec terrible pour notre société, qui ne peut faire vivre un véritable service public en la matière. c'est la recherche d'un nouveau territoire pour le marché ... Les rapporteurs de la commission des lois ne s'y trompent pas, puisqu'ils rappellent « la nécessité de concilier, par exemple, l'objectif d'encadrement de la sous-traitance avec le respect du principe constitutionnel de liberté, de concurrence et de l'industrie ». Nous n'acceptons pas que des missions régaliennes de sécurité soient confiées à des entreprises privées, aux contours mal définis, du fait de cette sous-traitance. Avec ce texte, le secteur de la sécurité privée se trouve doté de nouvelles compétences : autorisation à détecter les drones et à conduire des missions de surveillance sur la voie publique en matière de lutte contre le terrorisme, en particulier. Il voit aussi ses prérogatives renforcées en matière de contrôles Pour ce qui est de cet article, qui concerne l'encadrement de la sous-traitance, nous regrettons que la limitation de celle-ci, votée par l'Assemblée nationale, à la réalisation de 50 % d'un contrat passé, ait été supprimée en commission. Si tout est fait pour assurer le développement de ce secteur, appelé à la rescousse pour l'organisation de grands événements à venir, rien n'est prévu pour améliorer, par exemple, le statut des agents, qui souffrent,

Ce secteur, en plein développement depuis des années, avec plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est pour autant fragile et instable. La logique marchande qui imprègne le secteur de la sécurité privée est pleinement contradictoire avec les missions de service public de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre l'article 7.

À l'heure de l'organisation des prochains grands événements, comme la Coupe du monde de rugby ou les jeux Olympiques, nous craignons le recours massif, voire abusif, à la sous-traitance en cascade dans le domaine de la sécurité. En 2015, dans le cadre d'une QPC, le Conseil constitutionnel avait rappelé que le législateur s'était fondé sur un motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens pour limiter les conditions d'exercice de la sécurité privée. Je suis surpris que nous ne considérions pas le développement de la sous-traitance comme un risque d'atteinte à cet intérêt général de protection de l'ordre public. Aussi, mon groupe souhaite la suppression de cet article.

pour explication de vote. Nous avons fait un choix différent de nos collègues qui se sont exprimés à l'instant. Comme eux, nous sommes contre l'intégration des entreprises de sécurité privée dans ce continuum de sécurité.

Sabine Van Heghe. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial de la proposition de loi, afin d'appliquer le régime dérogatoire au régime général de la sous-traitance à l'ensemble du secteur de la sécurité privée, c'est-à-dire aux activités privées de surveillance, de gardiennage et de protection physique des personnes,

de la commission ? Nos collègues souhaitent que les règles relatives à la sous-traitance s'appliquent à toutes les entreprises de sécurité privée, alors que l'Assemblée nationale en a restreint le champ d'application aux entreprises de surveillance humaine et de gardiennage. matière de sous-traitance en cascade concernent uniquement ces entreprises, ce qui explique le fait le choix fait par l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que les entreprises visées assurent 70 % du chiffre d'affaires de l'ensemble de la sécurité privée. Ainsi, je ne crois pas qu'il soit utile d'étendre aux secteurs qui fonctionnent de manière saine, à savoir le transport de fonds, la surveillance électronique ou les gardes du corps, les contraintes importantes conçues pour moraliser le secteur de la surveillance humaine et du gardiennage. Veillons à ne pas surréglementer et surcontrôler lorsque la situation sur le terrain ne le justifie pas.

vise à poser des règles plus restrictives en matière de sous-traitance, mais son adoption aurait, en fait, le résultat inverse de celui qui est recherché, car elle supprimerait la limitation à deux rangs de sous-traitance, ainsi que l'obligation de justifier auprès de l'entrepreneur principal le recours à la sous-traitance. Avec la sous-traitance serait limitée à un tiers du travail, sauf si le donneur d'ordre donne son accord pour aller au-delà, mais cette référence au travail est floue : faut-il prendre en compte le nombre d'heures de travail ou le chiffre d'affaires réalisé ? Cela pose un problème de définition.

On l'a bien compris, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, l'ensemble des dispositions relatives à l'élargissement des possibilités d'intervention de la sécurité privée est censée

si l'on refuse de décliner la sous-traitance au deuxième degré ou si l'on veut limiter la sous-traitance à 50 %, c'est parce que l'on sait pertinemment que, à un moment donné, il sera très difficile de savoir quelles sont les personnes

veillé à professionnaliser, à sécuriser et à réguler le champ de la sécurité privée, qui est aujourd'hui une réalité dans notre pays. Encore une

prendre en compte les réalités et la faisabilité. Effectivement, il y a eu beaucoup de discussions autour de la délégation à des sous-traitants de second rang. Cela semble facile à faire, à partir d'un pourcentage de marché, mais je pense que c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, la sécurité privée est cantonnée à un champ d'intervention bien précis, et le métier est régulé. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'améliorer

qui devraient se conformer aux dispositions de l'article 7 au cours du même délai. À défaut, ce dispositif perdrait l'essentiel de son intérêt. Quel est l'avis de la commission ? de la commission ? Cet amendement est contraire à la position de la commission. Pour ne pas déstabiliser les relations contractuelles existantes, nous avons souhaité que les règles nouvelles relatives à la sous-traitance s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur. Les relations contractuelles évoluent en permanence au gré des mutations économiques. À moyen terme, il ne fait donc guère de doute que les nouvelles règles relatives à la sous-traitance s'appliqueront à la grande majorité des activités de surveillance et de gardiennage. Cependant, nous ne voulons pas obliger les donneurs d'ordre à remettre en cause, dans l'année qui vient, les relations contractuelles qui leur donnent peut-être

Toutefois, l'article 8, qui élargit les missions des agents de sécurité privée pour leur permettre de relever l'identité et l'adresse des auteurs présumés d'une infraction lors d'un contrôle, n'est pas soutenable. Nous nous opposons à la rétention d'une personne contre son gré par des agents de sécurité privée pour attendre l'arrivée d'un agent de la police nationale. Nous y sommes d'autant plus opposés qu'aucune durée maximale n'est précisée.

missions particulières de la police nationale, au profit des agents de sécurité privée. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons la suppression de l'article 8. La parole l'amendement n° 144 rectifié. Les prérogatives déjà attribuées aux agents de sécurité privée nous paraissent très importantes. La rédaction de certains procès-verbaux ou le relevé de l'identité doivent demeurer une prérogative de la police et de la gendarmerie. Les responsabilités de la police judiciaire sont en effet couplées à une formation adaptée et à une responsabilité renforcée. Certes, le rapporteur de notre commission a noté « avec intérêt la déclaration de bonnes intentions que constitue l'engagement du directeur du Cnaps de mettre en place un parcours d'habilitation et de formation pour garantir la qualité des procès-verbaux », ajoutant que « cet effort de formation conditionn[ait] la réussite de la réforme.

le citoyen mis en cause, qui ne souhaiterait pas s'y soumettre, devant, le temps que l'agent de sécurité prévienne un officier de police judiciaire, ou OPJ, pour effectuer ce relevé, rester à la disposition de l'agent du Cnaps, sous peine d'une sanction de deux mois d'emprisonnement.

de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continuellement garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes », à savoir les agents de sécurité privée, « par les officiers de police judiciaire ». Il conclut ainsi : « Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article XII de la Déclaration de 1789. Or, actuellement, il n'y a absolument pas de contrôle par les OPJ, qui ne sont pas présents ou qui sont très éloignés. Les risques d'abus, notamment lors de manifestations sociales, étant bien trop importants, notre groupe propose une suppression de cet article.

de veiller au respect de la réglementation applicable aux agents de sécurité privée, en particulier de lutter contre le travail illégal. Chers collègues, je ne comprends pas pourquoi vous proposez la suppression d'un tel article, car cela priverait ces agents de ces compétences, qui sont très utiles dans le cadre de la régulation de la profession.

ou d'assermentation aux agents de sécurité privée, mais de donner des pouvoirs supplémentaires aux agents publics que sont les agents du Cnaps,

la professionnalisation des agents de sécurité privée, la responsabilité découlant des pouvoirs qu'ils ont et la traçabilité de leur action- après tout, ils sont dans le continuum de sécurité, et nous les assumons comme tels -, ne soient pas perçues à la légère. J'invite vraiment le Sénat, monsieur le rapporteur, à reconsidérer sa position, parce que, s'il n'y avait pas cette sanction, l'interdiction ne serait reliée à rien,

de la commission ? La commission n'a pas été convaincue par la nécessité de créer une sanction pécuniaire spécifique qui pourrait être infligée par le Cnaps à des salariés en cas de manquement à leurs obligations professionnelles et déontologiques. Je vais vous expliquer pourquoi. de sécurité privée sont des salariés comme les autres. Ils peuvent être sanctionnés par leur employeur en cas de faute et éventuellement licenciés. Ils peuvent, par ailleurs, être sanctionnés par le Cnaps, qui peut prononcer une interdiction temporaire d'exercice, ce qui revient, d'ailleurs, à leur infliger une sanction pécuniaire. Ils peuvent, enfin, faire l'objet de poursuites pénales s'ils sont embauchés sans disposer de la carte professionnelle. De plus, je veux insister sur le montant de la sanction administrative, à savoir 150 000 euros, qui nous est apparue comme démesurée au regard des revenus de ces agents de sécurité privée. L'amendement proposé par le Gouvernement constitue un progrès, puisqu'il tend à ramener la sanction encourue à 30 000 euros, ce qui représente tout de même deux ans de salaires nets pour un salarié payé au SMIC et le double de l'amende prévue en cas de condamnation pénale. On se demande quels manquements pourraient justifier une pénalité financière si lourde, et, par comparaison, dans quels métiers

à condition, premièrement, que la définition de l'infraction ne soit pas exactement la même, et, deuxièmement, que l'échelle de la sanction administrative ne soit pas disproportionnée au regard de la sanction pénale. Je n'avais pas pris conscience que les montants envisagés,

pour contrôler la validité des autorisations d'entreprises de sécurité privée et des titres individuels d'agent de sécurité. Au-delà de la publication sur le site internet des décisions, cette base de données doit être mise à jour des décisions du Cnaps affectant les autorisations d'exercice et les titres individuels. L'objet du présent amendement est d'offrir aux acteurs du secteur un accès facilité aux décisions prises par le Cnaps sur les autorisations d'exercice et sur les titres individuels.

Le portail de téléservices permet d'effectuer des demandes en ligne, par exemple pour obtenir une carte professionnelle ; il permet de vérifier la validité d'une carte, d'une autorisation ou d'un agrément. Il est donc nécessairement mis à jour en permanence. Si une entreprise fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer, cette sanction sera consultable sur le portail.

nommer et de dénoncer. Il s'agit de faire connaître à un large public, et notamment aux potentiels clients, les sanctions les plus graves prononcées par le Cnaps. Pour atteindre cet objectif, la publication doit intervenir sur des supports grand public, à commencer par le site du Cnaps, mais aussi

en posant une telle condition en matière d'emploi, exigible aux seuls étrangers, ces modifications sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur la nationalité, contraire au droit international.

d'équilibre : elle a prévu que les ressortissants étrangers, hors Union européenne, devront justifier de trois années de séjour régulier sur le territoire national pour pouvoir prétendre à une carte professionnelle. Cette durée de trois ans nous paraît concilier efficacement deux impératifs : disposer d'un peu de recul pour apprécier les antécédents judiciaires du candidat, mais aussi ne pas fermer pendant trop longtemps l'accès aux métiers de la sécurité aux ressortissants étrangers, qui trouvent souvent

la jurisprudence serait alors identique sur l'ensemble du territoire national, ce qui me paraît être de bonne politique.

Tout mécanisme automatique poserait des difficultés. Je ne méconnais pas les difficultés que vous évoquez, monsieur le ministre, mais elles sont le lot commun de toutes les juridictions sur le territoire national. On sait ainsi que l'on ne juge pas de la même manière à Marseille ou à Tourcoing,

Borchio Fontimp. Les personnes qui souhaitent exercer des missions de sécurité privée ne peuvent décemment être connues des services pour des actes de rébellion ou d'outrage aux forces de l'ordre. Cet amendement vise donc à corriger cette incohérence. Il est en effet impensable pour nos forces de l'ordre que des agents de sécurité privée puissent avoir été condamnés pour des actes répréhensibles à leur égard. Plus qu'une interdiction de bon sens, cet amendement tend à imposer une juste limite à l'accès aux missions de sécurité, publique ou privée. Quel est l'avis de la commission ? dans la loi une liste d'infractions incompatibles avec l'exercice des métiers de la sécurité privée. Elle a préféré conserver le système actuel, qui laisse au Cnaps le soin d'apprécier si l'infraction

issue de la commission des lois, réduit la durée de détention d'un titre de séjour de cinq ans à trois ans pour les ressortissants étrangers souhaitant exercer une fonction de sécurité privée. privée. Elle supprime également la condition imposée aux ressortissants étrangers souhaitant exercer cette activité de surveillance de justifier d'une connaissance des valeurs de la République,

Si la commission des lois a tenté, par ces nouvelles dispositions, d'améliorer le texte, ces dernières ne sont, pour autant, pas acceptables pour nous. Le présent amendement a pour objet de supprimer le conditionnement de la délivrance de la carte professionnelle d'agent

superfétatoire à l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. L'amendement

contraire aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux, à la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail. » Pour résumer notre état d'esprit,

que le souligne la Défenseure des droits, « en posant une telle condition en matière d'emploi, exigible des seuls étrangers, ces modifications législatives sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur la nationalité contraire aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux, à la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail ». D'autre part, les fonctions de sécurité privée sont l'un des vecteurs d'intégration des étrangers sur le marché du travail français. Une durée de deux ans semble, dès lors, suffisante et, surtout, proportionnée à l'objectif.

jeunes agents, qui sont amenés à avoir des contacts avec le grand public et avec des autorités, soient en mesure de maîtriser les rudiments des principes de notre fonctionnement républicain.

quand une partie des missions consiste à rester derrière un écran et visionner des images ou à faire du gardiennage statique ? J'ai déposé

pour que la convergence des luttes soit parfaite, je retire mon amendement

: La parole est à M. Serge Babary. Cet amendement vise à assouplir le principe d'exclusivité prévu par l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure applicable aux activités de surveillance, afin d'autoriser les entreprises de sécurité privée

En effet, le cadre d'intervention des sociétés de surveillance est pour l'instant strictement limité aux atteintes à la personne et à la surveillance ou au gardiennage. Ces sociétés ne peuvent donc proposer d'activités accessoires. Élargir le champ d'activité des intervenants sécuritaires à des prestations d'assistance aux personnes à domicile permettrait de renforcer le secteur de l'intervention sur alarme et de soulager les SDIS, déjà particulièrement sollicités. de la commission ? Par cet amendement, il est prévu que les entreprises de surveillance humaine et de gardiennage, ainsi que les entreprises qui gèrent des systèmes de surveillance électronique puissent proposer toute prestation de service en lien avec leur activité principale de surveillance.

- afin de « rentabiliser » davantage la plateforme qui gère les alertes, en autorisant les salariés à répondre à des demandes variées : venir en aide à une personne âgée qui a du mal à se relever, mais aussi, pourquoi pas, intervenir en appelant un plombier, en cas de fuite d'eau, ou un chauffagiste, si la chaudière tombe en panne.

à l'encontre d'agents de la police et de la gendarmerie nationales se comprend et se justifie par le fait qu'ils exercent des missions de sécurité publique,

Légalement, certaines garanties existent déjà : le code pénal prévoit plus d'une dizaine de circonstances aggravantes pouvant s'appliquer à l'ensemble des faits de violence, notamment à l'encontre des personnes particulièrement exposées exposées aux faits de délinquance. De plus, rappelons qu'à la différence des agents de sécurité publique les agents de sécurité privée ne sont pas investis de prérogatives de puissance publique, ni en général de pouvoirs de police. La sécurité privée ne doit pas être considérée comme un prolongement du service public. Il n'est donc pas justifié que les agents de ces services puissent bénéficier des mêmes circonstances aggravantes que les agents publics. Par conséquent, le groupe Écologiste -Solidarité et Territoires demande la suppression du présent article.

Les représentants des salariés de la sécurité privée jugent la mesure opportune. Sur le fond, je ne crois pas que la création de cette circonstance aggravante puisse entraîner une confusion entre agents de sécurité privée, d'une part,

doivent figurer sur les tenues des agents privés de sécurité. Cet article vise à renforcer le sentiment d'appartenance des salariés à leur profession, en prévoyant que leur tenue comportera, en plus du logo de leur entreprise, des éléments d'identification communs. Il s'agit d'accorder à ces salariés une forme de reconnaissance symbolique.

qu'« elles se sont inquiétées, plus généralement, de la tendance consistant à confier aux salariés de la sécurité privée des missions plus étendues de surveillance de la voie publique, au risque d'entraîner une confusion avec les responsabilités qui incombent aux forces de l'ordre ».

renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui permet aux agents de surveillance et de gardiennage d'exercer leurs missions dans les périmètres de protection créés par cette même loi. Au sein desdits périmètres, ces agents peuvent assister les membres de la force publique afin de réaliser des inspections et fouilles de bagages, ainsi que des palpations de sécurité, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.

Dans ce contexte, l'association des forces privées de sécurité déjà sur place, et donc opérationnelles, offrirait une opportunité pour accomplir des missions de surveillance ou lever un doute. Leur intervention serait très encadrée et soumise à l'autorisation exceptionnelle du préfet pour assurer la constitutionnalité du dispositif. Il n'en demeure pas moins que la lutte contre le terrorisme est au coeur des missions régaliennes de l'État et qu'elle ne peut pas être déléguée au secteur privé, même dans ce cadre très restreint. L'article 14 place sur le même plan la lutte contre les vols, les dégradations et les effractions et la lutte contre les actes de terrorisme qui est pourtant un champ de compétences très particulier et d'action exclusive de l'État, de ses services de renseignement, de la police et de la gendarmerie nationales. En outre, cette mesure entretient la confusion entre les missions des forces de l'ordre régaliennes et celles, nécessairement plus limitées, dévolues aux agents privés de sécurité. Les forces de sécurité intérieure doivent conserver le monopole de la surveillance générale de la voie publique. L'inscription de cette autorisation dans la loi ouvre la voie à de possibles dérives sur les missions régaliennes.

L'article 14 de cette proposition de loi que vous proposez de supprimer, mes chers collègues, autorise les agents de surveillance et de gardiennage à exercer sur la voie publique, à titre exceptionnel et sur autorisation du préfet, des missions de surveillance contre les actes de terrorisme.

Il s'agit simplement d'autoriser la surveillance des abords immédiats d'un bâtiment- concrètement, en faire le tour. À la demande du client, l'agent de sécurité sera autorisé à surveiller ce qui se déroule à proximité immédiate du lieu dont il a la garde- sur le trottoir ou le parking -de manière à appeler l'attention des forces de l'ordre, s'il aperçoit par exemple une personne armée ou un colis suspect. Il ne s'agit évidemment pas de demander aux agents de sécurité de se substituer aux forces de police ou de gendarmerie dans la lutte antiterroriste, mais simplement de prolonger la mission de surveillance au-delà

ponctuelle et contrôlée. Il serait surprenant de la refuser dans le cadre d'une menace terroriste identifiée, alors qu'elle est permise en cas de risque d'effraction ou de dégradation. Alors que l'actualité nous montre régulièrement que la menace terroriste demeure élevée,

à des palpations de sécurité. Les palpations de sécurité ne sont pas des actes simples. Elles nécessitent une formation- le rapport de la commission souligne d'ailleurs que celle-ci est inégale. Elles portent atteinte à l'intimité des personnes. De plus, elles interviennent dans un contexte qui peut être tendu, voire dangereux. Il est donc de bon sens que le représentant de l'État garantisse aux personnes présentes, aussi bien qu'aux agents, un niveau de sécurité et de protection minimal. L'argument de la réduction d'une charge de travail non négligeable pour le Cnaps ne tient pas,

le secteur de la sécurité privée est extrêmement morcelé, avec un taux d'entreprises unipersonnelles très élevé, un fort turn-over, unrecours fréquent aux CDD, ainsi qu'une habitude de sous-traitance en cascade- nous en avons parlé lors de l'examen de l'article 7. De plus, la multiplication des domaines d'intervention et le contexte sécuritaire nous invitent à mettre en place un encadrement particulièrement strict et un suivi rigoureux. Avec quinze mille agréments donnés chaque année, le nombre d'agents habilités atteint des sommets et il faut pouvoir garder leur trace.

nécessaire à la garantie des droits. Aussi, le groupe Écologiste -Solidarité et Territoires souhaite la suppression de cet article pour en rester,, à un système d'habilitation.

du domicile. Les entreprises de télésurveillance pourraient, dans le prolongement des prestations qu'elles offrent au domicile, avec les mêmes garanties de qualité et sans aucune difficulté d'ordre technique, proposer à leurs clients d'utiliser leur smartphone un bouton d'alarme dans une situation de danger, et ce quelle qu'en soit la raison.

hors du cadre domestique serait strictement limitée à la détection à distance et à la mise en relation avec les forces de l'ordre ou les services de secours. Elle n'est envisagée que dans un cadre strict pour les entreprises concernées et sans intervention physique sur la voie publique. En outre, aucun enregistrement de son ou d'image ne sera possible, ni directement par le télésurveilleur, ni indirectement par l'intermédiaire de la personne protégée. Seul l'échange

amendement a pour objet d'autoriser l'extension des activités de surveillance à distance à la protection des personnes hors de leur domicile. L'intérêt pour la personne protégée, qu'elle soit âgée, vulnérable, seule, menacée ou accidentée,

ses clients. Lorsqu'une alarme se déclenche chez un client, une plateforme de surveillance reçoit une alerte et les salariés de l'entreprise effectuent une levée de doute. S'il apparaît qu'une infraction a été commise, ils appellent les forces de l'ordre pour qu'elles interviennent au domicile du client. L'idée serait d'étendre le service offert afin que le client, quand il quitte son domicile, puisse déclencher une alerte en cas de malaise ou d'agression,

aussi sur la valeur ajoutée d'un tel service. En cas d'agression, ne vaut-il pas mieux composer le 17 pour la police ou le 15 pour les secours ? L'intervention de la plateforme d'entreprise ne va-t-elle pas faire perdre un temps précieux ? Ces amendements

À la différence des agents de sécurité privée, les agents de sécurité incendie ne relèvent pas, actuellement, du livre VI du code de la sécurité intérieure.

En pratique, ces salariés sont amenés à intervenir dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur, parfois seuls et de nuit. Ils assument des missions essentielles pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il est donc légitime de s'interroger sur le bien-fondé d'une évolution de la législation dans ce domaine pour soumettre les professionnels de la sécurité incendie aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure. Tel est l'objet de cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Défavorable.